Cet amendement ne serait alors en discussion commune qu'avec les amendements incompatibles qui le précèdent dans le dérouleur. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé.

vers vous pour vous dire que nous aurons besoin, très rapidement au cours de ce débat, des réponses à ces deux problématiques. La première

jaunes. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe devant nos assemblées et dans toutes les villes de notre pays. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne et se mérite. Les Français qui s'interrogent ne sont pas tous des « antivax » ou des complotistes. Si les Français sont la plupart du temps opposés à vos mesures sanitaires, c'est que depuis le début de cette crise, nous avons entendu des discours confus et idéologiques, voire contradictoires

En plein état d'urgence sécuritaire, on nous explique que la Constitution et les libertés passeront toujours avant la menace terroriste. Aujourd'hui, on limite encore un peu plus la liberté des Français. C'est une évidence : le passe sanitaire opérera un changement majeur de notre modèle de société.

Je ne vous cache pas que, à l'image de nombreux Français, je reste très inquiète face à ce projet de loi, dont le dispositif soulève des questions à la fois éthiques et juridiques. Je crois en la responsabilité des Français

Je salue donc la rédaction de l'article 1 telle que l'a proposée le rapporteur de la commission des lois, Philippe Bas, dont la pertinence ne surprendra personne, ici. aura la faculté d'adapter l'état d'urgence sanitaire et d'y mettre fin selon la situation dans les territoires, elle satisfait un amendement que je projetais de déposer pour Saint-Barthélemy. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer pour vous demander d'emblée, madame la ministre, que ces modalités trouvent à s'y appliquer. En effet, l'accès à l'île est déjà conditionné à un contrôle sanitaire aux frontières, aussi bien pour la population que pour la clientèle touristique, cette dernière étant en très large partie vaccinée. Pour venir à Saint-Barthélemy, être vacciné ne dispense pas de réaliser un test PCR ou antigénique, mais seulement de rester une semaine à l'isolement à l'arrivée. Il y a donc, de ce point de vue, une double vérification.

À cet égard, notre clientèle touristique étant essentiellement américaine, pouvez-vous, madame la ministre, m'indiquer les modalités d'application du passe sanitaire pour les étrangers ? Aussi, bien qu'étant favorable à la vaccination, je suis opposée à l'extension du passe sanitaire à Saint-Barthélemy. C'est aussi la position du président de la collectivité, qui y est farouchement opposé, notamment pour les raisons que je viens d'exposer.

Protéger la population reste l'une de mes priorités, mais de nombreuses interrogations persistent sur les choix qui ont été appliqués dans mon territoire en matière de politique vaccinale.

a encore été récemment confirmée par les autorités sanitaires de l'archipel pour les tranches d'âge concernées et en fonction des critères qui étaient les vôtres. J'en appelle donc à la sagesse du Gouvernement, afin de mettre en place en urgence des mesures d'accompagnement des élus locaux

Ligne rouge », « anticonstitutionnalité », « Loïc, tu es un paranoïaque, qui voit le mal partout », « c'est impossible ! » ... Moins de deux mois plus tard, nous y sommes : le passe sanitaire est en voie d'être généralisé dans notre pays

du quotidien, ont donc changé d'avis et décidé de soumettre au Parlement un texte dans l'urgence et la précipitation, nous imposant- je le rappelle -des conditions d'examen épouvantables.

vaccinale pour tous, qui ne dit pas son nom. Les individus se feront vacciner, non pas pour contribuer au bien commun, selon une vision altruiste et fraternelle de la vaccination, mais parce que cela favorise les intérêts de chacun. Pire encore, avec ce passe sanitaire, nous nous apprêtons à entrer dans une société où le contrôle social de tous sur tous sera rendu possible, ce qui, encore une fois, est

dans l'édifice consolidé des motifs de licenciement et ouvre la boîte de Pandore à tout type de licenciement pour des motifs bien contestables. La commission des lois est revenue à la marge sur le dispositif proposé par le Gouvernement, mais celui-ci sera sans doute rétabli, ne nous leurrons pas. À l'inverse de ce type de mesures gravissimes pour nos libertés publiques, en totale rupture avec nos principes républicains, nous prônons, pour notre part, la pédagogie et l'information.

au bas des tours, au plus près de la population : ce seront 205 vaccinations dans la journée, dont 184 primo-vaccinations.

! Et c'est très bien ! Ce que vous nous proposez, c'est tout à fait autre chose. Je pense à cette femme de 80 ans que j'ai rencontrée dans un immeuble et qui ne veut pas se faire vacciner.

très concrètement ? Encore une fois, notre pays est en retard sur les événements. Nous étions en retard sur les tests, sur le gel, sur les masques, sur les vaccins. La campagne de vaccination, à partir du mois de janvier, a été chaotique. Aujourd'hui nous sommes également en retard sur le variant

fait. Notre solution, vous l'avez compris, ce n'est pas le passe sanitaire, nous nous y opposons. Notre solution, c'est la vaccination universelle, la vaccination obligatoire pour l'ensemble des Français qui relèvent de cette possibilité. M. Véran a indiqué hier que 12 millions de personnes

que les mouvements « antivax » et les mouvements populistes divers et variés s'engouffreront dans les interstices laissés par votre proposition gouvernementale. Nous le regrettons, et nous formulerons d'autres propositions dans quelques instants.

formuler des propositions alternatives qui étaient soutenues par les soignants et par des collectifs des hôpitaux. Deux mois plus tard, où en sommes-nous ? Certes, le virus et les variants sont retors, mais plusieurs plusieurs scientifiques alertaient déjà sur cette quatrième vague. Ce manque d'anticipation existe depuis le début de cette pandémie et contribue, conséquence de nombreuses volte-face, à créer colère, désespérance, mise en doute de la

dans une autre dimension, celle d'une société de contrôle et d'exclusion. Certes, on peut changer d'avis à la lumière de l'évolution d'une situation, mais avouez que cette rupture inédite est dangereuse. En effet, même si ce passe sanitaire est, pour vous, une incitation à la protection, dans les faits, vous provoquez de graves fractures. Alors que les mesures de restriction

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour nous, ce texte crée une brèche inacceptable dans le droit du travail. L'instauration du passe sanitaire dans les établissements recevant du public (ERP) va être imposée non seulement aux clients et aux usagers du service public, mais aussi aux salariés.

même ceux qui rendent la vie supportable- je pense notamment à tous les moments culturels. Il réduit la liberté de circuler, quoi que vous en disiez.

Nous savons que la carte du plus faible taux de vaccination recoupe celle de la pauvreté, de la fracture numérique, de l'accès au service public. C'est la Défenseure des droits qui le dit. L'extension du passe sanitaire ne fera qu'accroître ces inégalités

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment de discuter de l'article relatif à l'extension du passe sanitaire, il me paraît opportun d'appeler votre attention sur ses conséquences pour les Français de l'étranger qui souhaitent revenir sur notre territoire. Trois problèmes se posent. Tout d'abord, un grand nombre de Français de l'étranger n'ont pas encore été vaccinés. Nous apprenons en ouvrant nos mails qu'un appel d'offres a été passé par le Quai d'Orsay pour accélérer et élargir la vaccination à l'étranger. C'est heureux. Cette semaine encore, j'ai été alerté notamment par nos élus des Français en Algérie ou encore en Iran : l'attente est plus que forte. L'urgence est là, mais je ne vois rien dans le droit en vigueur ou dans les dispositions dont nous débattons qui garantisse Ensuite, il est nécessaire que les vaccins reçus par les Français établis hors de France dans leur pays de résidence leur donnent accès au passe sanitaire. Or, d'une part, le certificat de vaccination reçu à l'étranger n'est souvent pas reconnu par le système français,

une nouvelle catégorie : les vaccinés non vaccinés. Pour eux, notre secrétaire d'État a déclaré que le Gouvernement étudiait la faisabilité de l'inoculation d'une troisième dose d'un vaccin homologué afin qu'ils puissent détenir un passe sanitaire. Nos compatriotes devront-ils avoir leur surdose ? Reste le dépistage. Là encore, rien ne garantit que les tests seront bien pris en charge, comme le prévoit une très vague instruction du directeur général de la santé, qui n'est pas appliquée.

pharmaciens ne semblent pas très au courant ! Serait-il possible de prendre une véritable mesure normative opposable afin d'acter la gratuité des tests pour les Français de l'étranger ? Car, à l'évidence, il ne s'agit pas de tests de confort. Le passe sanitaire, tout comme l'enfer, est pavé de bonnes intentions. N'oublions pas non plus que l'enfer est dans les détails : ne faites pas de ce passe sanitaire un enfer pour les Français de l'étranger. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les interpellations ayant été assez nombreuses et fournies et les sujets abordés

à évoluer. J'en viens au point particulier de l'anticipation et je tiens à expliquer pourquoi, alors même que nous nous félicitions il y a quelques semaines du fait que l'épidémie était maîtrisée, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une forme de situation d'urgence.

Si nous voulions une approche beaucoup plus systématique, au vu des réserves émises par la CNIL sur l'accès au fichier des patients à risque Pardon, madame la sénatrice, mais je considère que le respect du Parlement consiste à répondre en détail à l'ensemble des questions qui ont été posées-sauf à ce que vous préfériez qu'il n'y ait pas de réponse ? On

n° 13 rectifié. Nous proposons la suppression de l'article 1, en cohérence et en coordination avec l'amendement que nous avons déposé et qui vise à instaurer une obligation vaccinale généralisée contre la covid-19, sauf contre-indications médicales, car ledit amendement prévoit une solution alternative au dispositif du passe sanitaire envisagé par le Gouvernement. Prenons le temps d'engager sereinement ce débat. Dans la perspective de l'examen du projet de loi de relatif à la gestion de la crise sanitaire, la commission des lois du Sénat a auditionné M. Olivier Véran le 22 juillet dernier. Interrogé sur l'obligation de vaccination universelle, le ministre a estimé que ce débat était légitime. Il a accueilli favorablement les propositions qui ont été présentées à ce sujet. Il a invité le Parlement à se saisir de cette question afin que puisse s'engager une discussion de fond à l'occasion de ce projet de loi, et il a assuré que le Gouvernement serait ouvert au dialogue. Sans mésestimer les améliorations apportées au dispositif proposé, nous restons opposés à cet article, qui procède au rétablissement du régime de l'état d'urgence sanitaire pour pour mieux valider l'élargissement du périmètre du passe sanitaire. Celui-ci, jusqu'à présent limité aux activités de loisir, foires ou salons professionnels, s'appliquera dorénavant à certaines activités quotidiennes comme la restauration, les débits de boissons, les voyages nationaux intérieurs, les centres commerciaux et les lieux d'accueil des publics vulnérables. De plus, tel qu'il ressort des délibérations de l'Assemblée nationale- et en dépit des modifications introduites par la commission des lois -, nous estimons que ce dispositif est inapplicable en pratique. Nous examinerons point par point Nous examinerons point par point le dispositif dans la rédaction adoptée par la commission des lois, pour en retirer les dispositions que nous jugeons inappropriées ou pour réintroduire celles qui nous paraissent nécessaires. En tout état de cause, qu'il soit clairement entendu que nous plaidons pour une extension généralisée et obligatoire de la campagne de vaccination contre la covid-19, seul chemin pour asseoir une immunité collective tout en assurant une égalité de traitement de la population, en particulier là où les inégalités territoriales et sociales d'accès à la vaccination sont les plus importantes. Seul ce choix vertueux nous permettra de sortir du dilemme dans lequel nous enferme le projet de loi : passe sanitaire et mesures d'isolement de plein droit en cas de contamination constatée, ou retour au confinement généralisé.

l'examen de cet article. Le choix de l'extension du passe sanitaire aux actes de la vie quotidienne des Françaises et des Français est révélateur d'une politique sanitaire axée sur la contrainte et la surveillance généralisées. Il impose un contrôle social de tous par tous et comporte un fort risque de fracture de notre société. Ce dispositif porte atteinte à notre État de droit sur de nombreux points. points. D'abord, imposer un passe sanitaire à tous les Français dans des délais qui ne leur permettront pas de se conformer aux nouvelles exigences est très problématique. C'est leur faire payer le défaut d'anticipation Sur le plan de l'accès aux données personnelles, le passe sanitaire généralisé impose de montrer un justificatif médical pour la grande majorité des actes de la vie quotidienne. Les données médicales et d'identité seraient ainsi consultables et consultées par tous, ce qui est contraire à l'éthique et à notre vivre-ensemble. Les commerçants, restaurateurs et personnes travaillant dans les activités de loisir n'ont pas pour mission de procéder à la surveillance de la population. Il y a ainsi de forts risques de troubles à l'ordre public car ces derniers, non formés à cette mission de contrôle, ne détiennent pas les pouvoirs de coercition de la police et de la gendarmerie. Ce contrôle s'avère, en outre, impossible à mettre en place en pratique. L'instauration d'un tel passe sanitaire présente, de fait, un véritable risque au regard des violations des libertés individuelles- liberté d'aller et venir, respect de la vie privée et familiale -et introduirait des ruptures d'égalité entre les citoyens. Les aménagements des rapporteurs en commission et l'instauration de deux régimes de passe sanitaire modulables en fonction de la situation sanitaire des différents territoires contribueraient à accroître l'illisibilité pour la population, qui déjà ne comprend qui déjà ne comprend plus guère les règles. Les Françaises et les Français ne pourront comprendre avec clarté des règles sanitaires applicables dans un territoire concerné par l'état d'urgence sanitaire et pas dans un autre, en régime de sortie. telle politique semble contre-productive, mais je n'ai pas le temps de développer ce point. Le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires dénonce avec force les nombreuses incohérences et le caractère liberticide de ces mesures. Il faut

du refus d'un programme de recherche en vue de trouver un traitement, ou encore du contrôle aux frontières. On préfère nous imposer de manière déguisée la solution unique de la vaccination obligatoire dès l'âge de 12 ans, sans possibilité de recours en cas d'effets secondaires, sans transparence sur la fabrication des vaccins, pas plus que sur les contrats aux montants pharaoniques qui en découlent. Le passe sanitaire, c'est la solution de facilité que vous avez trouvée face à une situation complexe. Vous nous mettez de force et collectivement le doigt dans l'engrenage de l'identification numérique, qui nous mène vers un régime inspiré par le Parti communiste chinois ! Quand on voit la puissance des menaces du cyberespionnage ces derniers jours, comment consentir à prendre de tels risques ? Nous refusons le piège du passe sanitaire. Les irresponsables, ce ne sont pas les Français qui usent de leur liberté, mais l'Union européenne, qui couvre les laboratoires en cas d'effets secondaires, secondaires, et nos dirigeants, qui font un chantage à l'obligation dissimulée derrière un passe sanitaire ultracontraignant. L'exemple d'Israël, sur le point de se résigner à un nouveau confinement, devrait offrir un vaccin d'humilité aux vaccinolâtres et aux donneurs de leçons 60 % des nouveaux contaminés en Israël sont vaccinés ! J'ai entendu le chef de la majorité de droite au Sénat, notre collègue Retailleau, dire que nous n'aurions le choix qu'entre le passe sanitaire et le confinement. Je suis persuadé qu'il se trompe, et je suis convaincu que nous aurons les deux : et le passe sanitaire, et le confinement. Exact ! Quant aux membres du Gouvernement, ils ont tous juré la main sur le coeur, il y a quelques semaines, qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Aujourd'hui, empreints de la même conviction, ils affirment le contraire Les mêmes qui se refusent à stigmatiser, ficher et traquer les ennemis de la France s'apprêtent à faire entrer de force la France tout entière dans un état de contrôle total, avec les discriminations et les restrictions de liberté qui en découlent. Il y a donc un laxisme à deux vitesses, et une fermeté à deux vitesses. Le Gouvernement a choisi ses ennemis ; la liberté, l'égalité et la fraternité sont confisquées. Par cet amendement, je m'oppose à toutes ces mesures de domestication étatique, pharmaceutique et « gafamique » imposées par ce texte. Nous n'acceptons ni de nous faire dicter notre comportement ... Merci de conclure

Quand on défend les libertés publiques, il faut accepter trois choses : être minoritaire, avoir raison trop tôt et mener un combat de long terme. Voter la suppression de l'article 1, c'est mettre un coup d'arrêt à cette fausse bonne idée qu'est le passe sanitaire et à son extension. Ce passe sanitaire pose des questions de principe considérables et des questions d'applicabilité qui ne sont pas moindres, comme cela a déjà été évoqué par un certain nombre de nos collègues. Pour certains, c'est un nouvel accommodement raisonnable, un nouveau mal nécessaire. Mes chers collègues, où cela nous emmène-t-il

de remettre en cause les engagements que vous avez pris ici même, au nom du Gouvernement, il y a seulement deux mois. Mes chers collègues, le passe sanitaire que nous votons aujourd'hui, nous risquons de l'avoir pendant des mois ou des années.

Au moment même où le ministre de l'intérieur écrit aux préfets pour leur dire que la situation est extrêmement périlleuse, que des menaces importantes pèsent sur la personne du Président de la République, sur lui-même, sur des responsables politiques, et que nous sommes dans une période où un attentat est peut-être imminent,

présenter l'amendement n° 168. Cet amendement vise à supprimer l'ensemble de l'article 1, dont les fondements reposent sur une volonté politique d'étendre de façon disproportionnée les contraintes liées à la détention du passe sanitaire, avec un risque de diviser et de fracturer bien plus encore notre pays déjà durement éprouvé depuis le début de la pandémie. Dans ce contexte de défiance généralisée, il convient de convaincre et non de contraindre. Or l'article prévoit d'organiser une société dans laquelle les citoyens se contrôleront les uns les autres et devront constamment justifier de leur état de santé sous peine d'amende. Je suis personnellement favorable à la vaccination, mais contre l'obligation, qui n'est qui n'est ni moralement, ni éthiquement, ni démocratiquement acceptable. En outre, cet article prévoit la prolongation du régime transitoire de sortie jusqu'au 31 décembre 2021, ainsi que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion,

Par exemple, une personne qui aurait enclenché le parcours vaccinal début juin et respecté le calendrier d'ouverture par âges pourrait se trouver exclue des lieux de vie sociale et culturelle en raison des délais entre les deux doses, et des sept jours d'attente pour obtenir son certificat une fois la seconde injection faite. C'est aberrant

que les TGV et les avions étaient les espaces les plus sûrs, tout en laissant une liberté totale dans le RER et métros bondés en Île-de-France ? Je ne vois là que de l'incohérence ... Finalement, vous faites porter la responsabilité de la gestion de cette crise à nos concitoyennes et concitoyens en les contraignant, en en les infantilisant. Mais quelle est la politique que vous menez pour combattre les inégalités sociales de santé ? Quelle politique conduisez-vous pour aller vers les populations qui habitent dans les territoires oubliés de la République ? Quels moyens développez-vous pour remettre à flot la médecine scolaire, ou la médecine du travail, qui est complètement mise à bas ? Voilà un certain nombre de questions auxquelles vous ne répondez pas ! Alors que nous sommes

Monsieur le président, on ne peut sans cesse opposer efficacité sanitaire et respect des libertés publiques. On ne peut pas avoir le respect absolu des libertés publiques dans le cadre de la sécurité sanitaire ; on ne peut pas régler la crise sanitaire sans admettre un changement de comportement qui exige une part de contrainte. Nous l'avons fait constamment depuis le début de la crise sanitaire. Puisqu'on ne peut pas opposer liberté et sécurité sanitaire, il faut réussir à les combiner. A-t-on trouvé la bonne mesure ? Nous, commission des lois, nous ne le pensons pas s'agissant du texte du Gouvernement, tel qu'il a été trop légèrement amendé par l'Assemblée nationale. Nous avons donc fait notre propre texte, en déplaçant

Et s'ils ont montré leurs limites, croyez-vous que du jour au lendemain, dans cette situation d'urgence, ces limites vont pouvoir être dépassées ? Pour ma part, je crois qu'il faut faire plus.

qui ne contamineront pas et ceux qui contamineront, un confinement : tous les Français à égalité ! Oui, nous Français, nous aimons l'égalité. Mais voulons-nous vraiment le confinement ?

» Oui, mais regardons comment dans les trois semaines qui viennent, c'est-à-dire au moment de cette flambée, on peut lui donner un coup d'arrêt par cette vaccination obligatoire. Si l'un d'entre vous a la recette

! Je ne sais pas comment, dans les prochaines semaines, nous pourrions arrêter la flambée de l'épidémie par la vaccination obligatoire. Cela ne disqualifie pas définitivement une mesure d'obligation pour la vaccination, certes, mais cela la rend impossible comme instrument alternatif à des mesures de freinage du développement de la crise sanitaire que nous connaissons depuis trois semaines.

utilisés jusqu'alors n'a été la martingale parfaite. Et ces martingales imparfaites ont tout de même fonctionné trois fois : le confinement, qui avait aussi des lignes de fuite, a pourtant permis de casser à trois reprises l'épidémie. Essayons donc de casser avec cette martingale imparfaite l'épidémie, avant de passer à autre chose s'il le fallait. J'espère bien que nous serons efficaces. Je ne crois pas

Ces règles, vous en êtes les dépositaires. Ce n'est pas par la peur du gendarme que nous vous demandons d'éviter la multiplication des contaminations, c'est par la conscience de votre responsabilité et de votre intérêt individuel à vous protéger.

la santé et le plus respectueux des droits individuels et des libertés. C'est tout le sens de la rédaction que nous avons adoptée. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de rejeter les amendements de suppression qui vous sont soumis.

je ne comprends toujours pas pourquoi les ministres de ce gouvernement ne veulent pas davantage travailler avec le Parlement. Mais bien sûr ! Je ne comprends toujours pas pourquoi, alors que nous traversons une crise sanitaire aussi dure pour tous, le Gouvernement a la prétention de tout savoir

Les contraintes et les restrictions liées au passe sanitaire ne sont pas des sanctions au sens juridique du terme. Ce sont des impossibilités de faire, des limitations de déplacement.

Si nous voulons inspirer confiance aux Français, il est temps de sortir de l'improvisation permanente et de marquer des lignes. Il faut affirmer que le vaccin protège et que la vaccination doit être universelle. Nous ne pouvons pas,

de perspective claire, nous ne pouvons être d'accord, monsieur le rapporteur, avec la philosophie dont vous nous avez fait part, qui est en totale cohérence avec celle du Gouvernement.

La plupart des sénateurs centristes voteront contre la suppression du passe sanitaire.

est-elle possible ? Oui probablement, à moyen terme, mais pas dans l'urgence. Plusieurs mois seront encore nécessaires.

Je voterai ces amendements de suppression. Je tiens à dire ici de manière lucide que je suis pour l'obligation vaccinale et contre le passe sanitaire tel qu'il nous est soumis, dans l'économie qui est la sienne. Je suis pour une vaccination obligatoire, planifiée,

et la liberté et la protection de la santé, qui est une exigence constitutionnelle, c'est l'obligation vaccinale. De même, je suis persuadé, contrairement à ceux qui disent

dernières années, démontre que la tendance est à la généralisation et à la pérennisation des mesures restrictives

Ce qui est sûr, monsieur le secrétaire d'État, c'est que vous n'avez pas été capables d'apaiser l'angoisse du peuple français. Pis, vous l'avez alimentée par vos déclarations contradictoires et vos prises de position successives.

Le scrutin est clos.

décembre 2021 une déclaration d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 octobre 2021. Cette déclaration généralisée n'apparaît pas adaptée à l'état de la situation sanitaire actuelle, qui, si elle montre des signes de reprise dans de nombreux territoires, ne présente pas toutes les caractéristiques d'une catastrophe sanitaire telle que celle que nous avons pu constater lors des déclarations précédentes. Le Gouvernement souhaite recourir à l'état d'urgence sanitaire exclusivement dans les territoires confrontés à des risques sanitaires d'une criticité particulière, en cohérence avec l'esprit du régime créé par le législateur en mars 2020. En outre, une nouvelle déclaration de l'état d'urgence sanitaire (EUS), dont le régime permet des interdictions ou des fermetures généralisées, serait contradictoire avec l'objectif du présent texte de développer des outils permettant de maintenir les différentes activités quotidiennes en les conciliant avec une maîtrise de la situation sanitaire, notamment l'extension du périmètre du passe sanitaire ou l'augmentation de la couverture vaccinale.

m'y refuse. Cela fait près de deux ans que nous vivons sous ce régime de restriction des libertés, toujours plus intrusif et élargi, pour le résultat que l'on connaît. Nous ne sommes plus dans l'urgence ; il faut penser les choix politiques à moyen et long terme. M. Delfraissy, président du conseil scientifique, a indiqué qu'un nouveau variant arriverait cet hiver, et que nous ne serions pas débarrassés du virus avant 2023. Il faut donc, enfin, nous organiser

relevait à la fois de la méthode Coué, du déni et d'une véritable provocation. Vous ne pouvez vous affranchir plus longtemps du contrôle parlementaire. En septembre, nous sommes à votre disposition pour réexaminer vos prérogatives. En continuant à nous imposer une pseudo-urgence, vous vous habituez au pouvoir total et aux restrictions de liberté sans protéger mieux les Français, sans prendre à bras-le-corps les problèmes structurels de notre système de santé. Combien de lits avez-vous ouverts depuis début 2020 ? Du 1 janvier au 31 mars 2021, en pleine pandémie, point d'ouvertures, mais 1 800 suppressions, si l'on en croit un syndicat infirmier. Par ailleurs, qui peut croire que l'état d'urgence ne sera pas encore repoussé après le 31 octobre ? Sans aucune réelle opposition parlementaire, mes chers collègues, je ne me fais que peu d'illusions. Par cette vision court-termiste, nous sommes en train d'hypothéquer notre avenir économique et social, au minimum pour la décennie à venir. À ce rythme, la prorogation sans fin de l'état d'urgence empiétera sur le bon fonctionnement démocratique puisque les restrictions de liberté entraveront le bon déroulement de la campagne présidentielle. L'abstention record des élections municipales, départementales et régionales devrait vous servir de leçon. Une urgence de deux ans, ce n'est plus une urgence, cela devient une permanence. Cette disposition constitutionnelle d'état d'urgence n'a plus lieu d'être ; nous sommes en train d'en galvauder l'esprit. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement de suppression de l'alinéa 3 et à refuser la prorogation de l'état d'urgence au-delà du 30 septembre. L'amendement

ne concernerait que la gestion de la crise sanitaire. Malheureusement, dix-huit mois après, nous y sommes encore ! Évidemment, l'épidémie se poursuit, mais, surtout, durant cet état d'urgence

et cela nous semble important. Nous ne soutenons pas la position du rapporteur, désormais adoptée par la commission des lois. Et puisque c'est le texte de cette dernière qui nous est soumis, nous souhaitons une intervention plus régulière du Parlement.

et solitaires. Nous devons gérer ces crises de manière plus durable et concertée. Le Parlement et la loi doivent jouer leur rôle plein et entier.

C'est une véritable remise en cause de notre modèle de société puisque, pour la première fois dans notre pays, les espaces publics, les actes du quotidien, les établissements recevant du public, les événements sportifs et culturels seront accessibles de manière différenciée aux citoyens français selon leur état de santé. Il s'agit d'un très grave recul de nos libertés publiques et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Une crise sanitaire ne peut devenir le prétexte à une remise en cause de nos principes fondamentaux, tels que l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la liberté. Ces principes fondamentaux sont essentiels pour garantir notre État de droit, y compris et surtout dans les moments de crise : il s'agit de garde-fous auxquels on ne doit pouvoir déroger. Il convient par ailleurs de souligner que les termes de ces textes sont particulièrement extensifs, laissant une grande marge d'interprétation au Gouvernement, avec des qualifications comme « activités de loisir » et « transport public de grande distance ». Voilà pourquoi je vous propose de supprimer ces dispositions, mes chers collègues.

La Guyane se distingue également par une mesure unique qui cristallise aujourd'hui le ressentiment de la population et qui ne se justifie plus depuis bien longtemps : l'instauration de frontières intérieures. Entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni vers l'ouest, ou entre Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock à l'est, vous devez franchir un barrage de police permanent, quel que soit le sens de circulation, et justifier votre passage par un motif impérieux.

Le constat est sévère car, lors de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, la Guyane n'était quasiment pas touchée, contrairement au reste du pays qui connaissait sa première vague. Celle-ci n'a atteint la Guyane que trois mois plus tard.

et de l'offre de services à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir pour l'heure à la vaccination. Monsieur le secrétaire d'État, il est urgent de prendre en considération les contraintes particulières de ces collectivités, dans la logique de différenciation que le Président de la République avait revendiquée pour les territoires français. L'amendement n°

La situation actuelle est la résultante des carences de l'État, des incohérences successives et de la volonté manifeste de diviser le pays. Il faut désormais éviter les conséquences systémiques. C'est la raison pour laquelle je vous présente cet amendement,

efficacement, en imposant des disciplines nouvelles. Enfin, l'état d'urgence n'implique évidemment pas de devoir recourir à d'autres moyens que ceux qui nous sont proposés. En particulier, si le Gouvernement devait décider le confinement ou des mesures de couvre-feu, il faudrait alors qu'au bout de trente jours, le Parlement les ait autorisés, selon le régime

on croit rêver par rapport à la situation que nous connaissons ! Si nous voulons que ces mesures, que nous pourrions adopter

nos outils de gestion de la crise sanitaire » ... Nous n'en sommes plus là ! Nous sommes en train de prendre des mesures extrêmement graves. Il faut dire la vérité, ne pas dramatiser, certes, mais ne pas sombrer dans l'euphémisme non plus.

qui a permis de lutter contre la crise sanitaire, et qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre de cette année. Je pense qu'il faut le conserver. Avis défavorable. Gontrie, même si vous avez pris beaucoup de précautions dans l'exposé des motifs de votre amendement, je comprends que, puisque vous voulez ramener du 31

de l'intensité de la circulation virale dans nos collectivités d'outre-mer, et du fait que la vaccination ne s'y propage qu'avec retard par rapport

Plusieurs collègues ont souhaité obtenir de la part du Gouvernement une forme d'engagement sur le respect du travail des commissions sénatoriales concernant l'article 1.

que ce que nous allons voter aujourd'hui. Je vous rappelle par exemple que, dans le cadre de l'article 16 de la Constitution, le Parlement se réunit de plein droit. Par ailleurs, sénateurs et députés peuvent demander au Conseil constitutionnel d'examiner les conditions qui justifient la prolongation des pouvoirs de crise, ce dont nous ne disposerons pas avec ce texte. donc un travail constitutionnel à mener. Je regrette vivement que le Gouvernement ait convoqué le Parlement pour une réforme constitutionnelle dont l'essentiel, de façon très artificielle,

Je pense que c'est un très mauvais signal donné à la Haute Assemblée, et je le regrette. explication de vote. Pour être très clair, je voterai contre l'amendement présenté par le Gouvernement, mais je soutiendrai les amendements présentés par le président Patient et par ma collègue Victoire Jasmin.

Au vu des contraintes historiques imposées aux Français, cela serait la moindre des choses. Dans un contexte de multiplication des variants du virus, il nous faut imposer, en plus de la fermeture des frontières aux clandestins, ce qui devrait être le cas en permanence, des contraintes sanitaires minimales pour entrer sur notre territoire. Malte, pays membre de l'Union européenne, avait mis en place ce protocole avant de le retirer, ce qui prouve que l'idée est fondée sur des craintes avérées face aux risques encourus. En ne votant pas cet amendement, mes chers collègues, vous renoncerez à régler le problème des variants, qui va devenir vous nous empêcherez, par ailleurs, de retrouver notre attractivité touristique. Je vous invite donc à adopter cet amendement de cohérence. Je précise que cet amendement a été porté par bon nombre de mes collègues députés du groupe Les Républicains. L'une des grandes constantes dans la gestion de l'épidémie par ce gouvernement a été l'absence de contrôle efficace de nos frontières. Compte tenu des contraintes accrues que le Gouvernement entend faire peser sur les Français dans les semaines à venir, il convient que notre pays se protège mieux des potentielles propagations de l'épidémie venant de l'extérieur, notamment dans un contexte de développement de variants. En fait, ce que je propose ici, c'est une mesure de cohérence. Nous allons imposer le vaccin à un certain nombre de personnes- je pense notamment aux professionnels de santé - ; on peut le comprendre et être pour. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous s'accordent sur

non seulement nous n'avons pas fermé les frontières avec l'Italie, mais, pire encore, c'est l'Italie qui a dû fermer les frontières avec la France. Aujourd'hui, alors que nous imposons le vaccin aux Français,

amendement est satisfait. Je vous recommande, ma chère collègue, de vous référer au 1° du III de l'article 1, tel que nous l'avons adopté en commission : vous constaterez par vous-même que ce contrôle aux frontières a bien été introduit. Par conséquent,

En 1720, le Comtat Venaissin a édifié un mur pour se prémunir de la peste qui venait de Marseille.

Selon nos informations, à ce jour, les mineurs n'auront pas besoin de passe sanitaire à l'école, mais devront en posséder un pour aller sur une base de loisirs. Cohérence, quand tu nous tiens ... Cette forme d'arbitraire dans vos décisions n'a aucun sens. la colère que l'on constate dans les manifestations successives. Elle exprime une fatigue, une lassitude face à ces nouvelles contraintes pour les libertés collectives, face au poids de ces nouvelles normes administratives, face à la déconnexion du pays légal par rapport aux pays réel. En effet, la loi ne fait plus sens quand on expose des enfants de 12 ans à des risques de myocardie, selon le président du Conseil national professionnel de pédiatrie, avec la vaccination, qui, elle-même ne leur apporte aucun bénéfice puisque ce virus ne les atteint pas dangereusement. Regardez vous-mêmes les statistiques des personnes décédées de cette maladie : en deçà de 45 ans, il n'y a déjà presque plus de risques. Sauf cas de comorbidités, bien sûr, aucun mineur ne meurt de ce virus. Or on ne vote pas une loi générale pour des exceptions. Alors, quel est le sens de cette disposition législative liberticide, qui est clairement disproportionnée ? La protection des données personnelles des mineurs et de leur vie privée doit être particulièrement garantie.

Parmi les très nombreux problèmes opérationnels de mise en oeuvre du passe sanitaire figure le choix d'imposer un passe sanitaire à des enfants : 12 ans, c'est l'âge de la cinquième, ayez bien cela en tête ! Je suis personnellement concerné, pour avoir des enfants de cet âge-là.

Je partage complètement l'argumentaire de M. Loïc Hervé, et je ne vais pas le répéter. Pour ma part, je veux pointer un problème de droit majeur, madame la ministre, sur lequel il faudra que vous nous répondiez. L'autorisation des deux parents est nécessaire pour permettre la vaccination d'un mineur. un mineur ne peut pas se faire vacciner sans la double autorisation de ses parents. Si vous le soumettez à un passe sanitaire,

de la Défenseure des droits, le 20 juillet dernier : « [ ...] l'accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

subordonner l'exercice de ce droit d'accès aux loisirs et au sport à l'obtention du passe sanitaire, sachant qu'un des deux parents peut s'opposer à la vaccination. Il y a là un point juridique lourd sur lequel nous souhaiterions absolument une explication. L'amendement

Il apparaît que l'âge de 15 ans est plus pertinent, car il correspond à l'entrée au lycée, qui coïncide bien souvent avec une augmentation des interactions sociales. Pour les collégiens, et plus généralement pour les mineurs de moins de 15 ans, les interactions sociales sont moindres et la mise en place du passe sanitaire pour cette catégorie de population semble disproportionnée.

Priorisons plutôt, et incitons à la vaccination des personnes vulnérables, des plus de 65 ans, des adultes en général ou des jeunes adultes de 15 à 18 ans, qui ont évidemment des liens sociaux plus importants que les jeunes enfants.

Je suis donc saisi d'une demande de la commission tendant à réserver l'examen de l'article 1 avant l'article 5. Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.